l'adjonction d'obligations supplémentaires ; l'extension du champ d'application de la directive ; la non-exploitation des possibilités de dérogations ouvertes par la directive ou le règlement, qui sera le cas à l'article 16 ; le maintien d'obligations antérieures à l'harmonisation européenne, ce qui était le cas hier soir à l'article 6. bien sûr, y avoir une combinaison de deux, voire de trois des définitions que je viens de donner. En deuxième lieu, je dois relever qu'il y a confusion entre mon rapport et le projet de loi.

revanche, le projet de loi que nous examinons n'est pas centré sur l'entreprise et son intitulé est clair

Ce texte traite de vingt-sept cas, qui relèvent de l'une au moins des définitions que je viens de donner. Il ne prétend pas traiter la totalité des surtranspositions. En troisième lieu, je rappelle que nous sommes au début d'un processus qu'il appartient au Sénat de poursuivre, de concert avec le Gouvernement.

J'ai également annoncé que le Sénat travaillera ensuite sur une proposition de loi de suppression d'une nouvelle série de surtranspositions, législatives cette fois.

J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que mettre le sabre au clair à la vue des vingt-sept suppressions proposées ne me paraît pas être le meilleur moyen de s'engager sur le long, difficile et politiquement périlleux chemin de la suppression d'un maximum de surtranspositions. Dans la

l'article 8, qui lui-même supprime l'obligation de consultation annuelle de l'assemblée générale des actionnaires en matière d'enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risques, prévue par l'article L. 511-73 du code monétaire et financier. monétaire et financier. Nous considérons que cette surtransposition se traduit par une formalité administrative peu contraignante pour les sociétés concernées, tout en garantissant, ce qui est, pour nous, très important, un degré d'information utile des actionnaires. Il y a donc lieu de supprimer l'article Quel est l'avis de la commission des dirigeants et preneurs de risques des établissements de crédit et des sociétés de financement. Cette obligation, qui n'est pas prévue par la directive, est clairement une surtransposition, et elle n'existe, j'y insiste, dans aucun autre pays européen. insiste, dans aucun autre pays européen. L'organisation d'une assemblée générale n'est pas, comme le considèrent les auteurs de cet amendement, une « formalité administrative peu contraignante ». Ce processus, fortement encadré, implique de réunir un quorum minimal d'actionnaires, parfois localisés à l'étranger. L'identification des personnes preneuses de risques et placées dans les fonctions ciblées peut être très complexe et demander un travail de recherche et de compilation fastidieux. Plus généralement, cette obligation pèse sur la capacité du secteur bancaire français à attirer des employés et administrateurs de qualité, susceptibles de contribuer au développement de la place financière de Paris. Ce signal est particulièrement dommageable au vu de l'enjeu que représente la relocalisation des établissements bancaires après le Brexit. L'avis de la commission spéciale est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'une

Dans le cas qui nous occupe, cette obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires ne trouve d'équivalent, cela a été dit, chez aucun de nos partenaires européens et introduit donc une distorsion de compétitivité avec ces derniers. ces derniers. Supprimer l'obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires porte-t-il atteinte au droit de regard de ceux-ci sur la politique de rémunération de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement ? Nullement. En effet, en vertu notamment de l'article L. 511-72 du code monétaire et financier, le conseil d'administration adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en oeuvre.

ne vois, dans le travail que nous essayons de faire, aucune remise en cause du principe de suppression des surtranspositions. Les interventions des uns et des autres, en prélude à l'examen de ce texte, étaient relativement unanimes sur cette question.

Toutefois, en l'absence des précisions apportées par le considérant 15 de la directive, l'ordonnance de 2016 ne retranscrit pas pleinement la volonté exprimée par le biais de la directive et ne permet pas de sécuriser la situation des opérateurs privés.

Cette jurisprudence met en évidence l'incertitude juridique. Il est clair, s'agissant des conventions de terminal, que leur requalification systématique en concessions serait un retour en arrière. Elle effacerait le progrès réalisé en matière de relance économique des ports français par la réforme portuaire de 2008. J'ai en ma possession une lettre de Philippe Juvin, député du Parlement européen et rapporteur du projet de directive. Il m'écrit L'intention du législateur, telle que précisée dans le considérant 15 de la directive Concession, est sans ambiguïté. Nous avons souhaité exclure du champ d'application de la directive les activités des opérateurs économiques exploitant les terminaux des ports maritimes ». J'ai également un courrier d'Alain Vidalies,

un cadre légal plus contraignant que celui qui est applicable dans les autres ports européens ou, plus généralement, inadapté pourrait désavantager les terminaux situés en France par rapport à leurs concurrents européens et internationaux. Dans cette fiche d'évaluation, il est demandé de légiférer

le port du Havre a lancé des appels à concession et l'on en est à attribuer les marchés. Autrement dit, un certain nombre de ports s'engouffrent dans cette faille juridique,

spéciale ? Cet amendement a pour objet de préciser le régime applicable en matière de contrat de concession pour les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports. suite du travail de la commission spéciale, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'une surtransposition en droit français : le cas visé par l'ordonnance reprend mot pour mot celui qui est prévu par la directive Concession.

collègues, nous comprenons qu'il s'agit d'un sujet important, dont plusieurs d'entre vous ont été saisis. Cela étant, la commission spéciale a proposé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement, afin de voir s'il partage ce constat et quelles perspectives il peut nous proposer.

que certains contrats d'occupation du domaine public soient requalifiés en concessions dès lors qu'ils ne se limitent pas à définir les modalités d'occupation du domaine public, mais qu'ils ont pour objet principal de répondre aux besoins de l'autorité concédante. Le Gouvernement partage l'objectif de clarté que vous recherchez, monsieur le sénateur Vaspart. Toutefois, le 2° de l'article 13 de l'ordonnance qu'il est proposé de modifier ne vise pas de telles situations. Il a pour objet d'exclure du champ d'application de l'ordonnance les contrats par lesquels les autorités concédantes acquièrent ou prennent en location pour leurs propres besoins des biens immobiliers, afin, par exemple, d'y installer leurs bureaux, et non les contrats de concession par lesquels une partie du domaine public est mise à la disposition d'opérateurs économiques. Afin de procéder à cette clarification, qui ne relève pas directement, comme l'a dit le rapporteur, d'une problématique de surtransposition, le Gouvernement a l'intention de proposer, dans le cadre du prochain projet de loi d'orientation d'orientation des mobilités, que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, des dispositions traitant spécifiquement de ce point, s'agissant en particulier des conventions d'exploitation de ports maritimes. En revanche, l'adoption du présent amendement ne permettrait pas d'atteindre l'objectif fixé. Son dispositif est, en tant que tel, dépourvu de portée juridique et, en tout état de cause, surabondant, dès lors qu'une mesure nationale de transposition est toujours interprétée par les juridictions à la lumière de la directive.

Le travail mené par la commission spéciale a fait apparaître que l'ordonnance de 2016 ayant transposé la directive de 2014 sur les concessions exclut de son champ d'application, et donc des règles relatives à la publicité et à la mise en concurrence qu'elle prévoit, les contrats de concession de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens. L'amendement examiné tend à préciser que ce régime d'exclusion est applicable « en particulier dans les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports

Le considérant de la directive Concession énonce que certains accords visant à exploiter certains domaines publics dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports ne devraient pas être qualifiés de contrats de concession. Or l'amendement tend à leur donner la qualification de concessions, certes exclues du champ de l'ordonnance de 2016, mais de concessions tout de même. Cela reviendrait donc à créer encore plus de confusion dans l'appréciation de la nature de ces contrats. L'avis de la commission spéciale

notamment comme des conventions d'occupation du domaine de l'ensemble des opérateurs des grands ports français. On est donc en train de faire fi de la loi de 2008.

de surcoûts. Sa suppression ne remettra pas en cause la protection de l'environnement et de la santé, parce qu'elle ne modifie pas les règles générales applicables à la gestion des déchets. à la gestion des déchets. Les opérations de gestion des déchets continueront d'être effectuées soit dans des installations classées, soit dans des installations de petite taille qui présentent suffisamment peu de risques pour l'environnement et la santé pour justifier de ne pas être classées. Ces installations non classées sont, par exemple, des installations de réparation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'image de ces objets du quotidien que sont les machines à laver, ou des installations de nettoyage de textiles gérées par l'économie sociale et solidaire. solidaire. Par ailleurs, les critères de sortie du statut de déchet sont issus d'une réglementation spécifique et fixés, au cas par cas, par un acte administratif, décret ou arrêté. Toutes les installations qui « feront » de la sortie de statut de déchet continueront donc d'y être soumises.

Ces modalités n'élèveraient pas le niveau de protection de l'environnement et de la santé, mais mettraient des freins supplémentaires au développement de l'économie circulaire, en particulier pour les acteurs les plus petits, comme ceux de l'économie sociale et solidaire. Pour ce qui est plus particulièrement des déchets dangereux, la plupart des installations étant classées dès le premier kilogramme de déchets traités, la levée de la restriction de la sortie du statut de déchet aux seules installations classées ne modifie pas, dans les faits, la situation actuelle.

La sortie du statut de déchet pour les déchets dangereux ne sera alors possible que dans les installations classées du type ICPE ou IOTA. Voilà qui me semble de nature à répondre aux préoccupations soulevées lors de l'examen du texte en commission, tout en évitant d'aboutir à la procédure actuelle pour les déchets non dangereux.

L'article 15 supprime, en droit français, la condition d'une valorisation uniquement dans une installation classée pour qu'un déchet cesse d'être un déchet. Cette suppression s'appuie sur l'argument selon lequel la directive prévoit bien la condition d'une valorisation pour cette procédure de sortie du statut de déchet, mais sans préciser qu'elle doit avoir lieu dans une installation classée. Premièrement, la même directive exige bien que, pour sortir du statut de déchet, les critères de la procédure doivent garantir un haut niveau de protection environnementale et prendre en compte des procédés et techniques autorisés, ce qui semble renvoyer à notre législation sur les installations classées. La surtransposition n'est donc pas, à mes yeux, caractérisée. Deuxièmement, la commission spéciale a estimé qu'il y avait un risque pour l'environnement et la santé humaine s'agissant des déchets dangereux, utilisés comme substituts de matière vierge dans des installations de production non obligatoirement classées. Pour cette raison, nous avons choisi d'assouplir le principe d'une procédure de sortie du statut de déchet exclusivement réservée aux installations de type ICPE, en prévoyant des dérogations possibles pour les déchets non dangereux.

La biodiversité disparaît à grande vitesse. Cela devrait nous mobiliser, nous conduire à nous interroger. Quelque 60 % des oiseaux sauvages ont disparu en quarante ans. Un tiers des oiseaux de nos campagnes ne sont plus, et cela en quinze ans seulement. Ce n'est pas rien ! À vrai dire, c'est d'ores et déjà un désastre. La menace est donc bien réelle et se précise de jour en jour, au fil des rapports qui se succèdent. La disparition des espèces vivantes sur Terre est en accélération. Au bout du bout, c'est nous qui sommes menacés. présent article va à l'encontre de tout ce que, ensemble, nous devrions mettre en oeuvre pour préserver le plus possible les espèces vivantes sur Terre. En effet, nous sommes dépendants de tout le vivant. Nos destins sont liés. Les rapports successifs appellent à des mesures radicales. Nous y sommes ! J'entends les arguments des uns et des autres : c'est trop tard. Au nom d'un intérêt supérieur, il y a notre responsabilité. Oui, il va falloir faire des sacrifices, d'autant que, s'agissant du présent article, il ne me semble pas que les dégâts soient tels que l'on soit obligé de légiférer. N'oublions pas que les oiseaux migrateurs vont subir eux aussi le réchauffement climatique et vont être fragilisés. C'est maintenant, les sacrifices ! Nous ne pouvons pas continuer comme avant. C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, de voter cet amendement, un pas sur le chemin vertueux de la préservation du vivant sur Terre. La

de certaines espèces d'oiseaux pendant les périodes de protection fixées par la directive Oiseaux. Alors que le projet de loi, cela a été dit à maintes reprises hier soir, énonce dès la première ligne de son exposé des motifs que l'excès de normes est pénalisant pour la compétitivité des entreprises,

avec l'objectif de rétablissement d'une concurrence plus loyale entre les États membres est en effet loin d'être évident, et ce d'autant moins qu'il n'y a pas de dégâts causés par les oies en

et il a été montré que les oies responsables de dommages agricoles dans les autres pays sont principalement issues de populations devenues sédentaires. Sur le fond, cet article revient en réalité à repousser la date de fermeture de la chasse des oies au-delà du 31 janvier. Cette mesure va à contre-courant de l'approche de la protection de la biodiversité encore réaffirmée au sein de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, ou dans le plan Biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà jugé en 2003 qu'une dérogation au titre de l'article 9 de la directive Oiseaux ne pouvait avoir pour véritable objectif de prolonger les dates de chasse. Nous sommes pourtant, en matière de

Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation du Sénat de Côte d'Ivoire conduite par son président, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio. À ses côtés se trouve André Reichardt, président du groupe d'amitié Afrique de l'Ouest. Je suis particulièrement heureuse de souhaiter à la Côte d'Ivoire la bienvenue dans la grande famille du bicamérisme, puisque ce pays a décidé d'instaurer un Sénat, à la suite de l'adoption de sa nouvelle Constitution, en novembre 2016. Dans le cadre de la mise en place du Sénat en Côte d'Ivoire à l'issue des élections sénatoriales du 25 mars 2018, un protocole de coopération parlementaire a été signé ce matin entre le président Gérard Larcher et le président Jeannot Ahoussou-Kouadio. Ce protocole, qui donnera lieu à des actions régulières de coopération sur différentes thématiques, sera mis en application dès demain. Les premiers échanges se tiendront avec des sénateurs et fonctionnaires du Sénat ivoirien. Ils porteront notamment sur le bicamérisme, sur la mission législative du Sénat, sur l'articulation entre le travail en commission et le travail en séance publique et sur l'organisation administrative et le fonctionnement du Sénat. En outre, la communication institutionnelle et les activités internationales du Sénat seront présentées à la délégation ivoirienne. La coopération entre les deux sénats devrait également s'intensifier dans les mois à venir, puisque le président du Sénat de Côte d'Ivoire a été convié à participer à l'Assemblée des sénats d'Europe, qui se tiendra, à Paris, du 13 au 15 juin 2019, sous la présidence du président Larcher. Pour la première fois dans l'histoire de cette assemblée, un dialogue sera en effet noué avec des secondes chambres africaines. Au nom du Sénat de la République française, je souhaite au président du Sénat de la République de Côte d'Ivoire et à sa délégation la plus cordiale bienvenue. Je forme des voeux pour que leur séjour en France soit profitable et contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux pays.

rectifié et 25 rectifié ? Ces trois amendements visent à supprimer l'article 16. Comme j'ai eu l'occasion de le dire devant la commission spéciale, cet article soulève un certain nombre d'interrogations quant à sa justification au sein de ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le débat puisse avoir lieu en séance publique sur le sujet. Mes interrogations sur cet article ont porté, premièrement, sur la plus-value apportée par celui-ci et deuxièmement, sur sa justification au sein de ce projet de loi de dé-surtransposition. Cet article complète l'article L. 424-2 du code de l'environnement qui fixe les règles du temps de chasse des oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, cet article du code précité détermine le principe d'une interdiction de chasser les oiseaux migrateurs, en application de la directive Oiseaux de 2009, pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Il comporte aussi une dérogation, prévue également par la directive pour les chasses traditionnelles, autorisant à chasser les oiseaux migrateurs en petite quantité et de manière strictement contrôlée et sélective. L'article 9 de la directive européenne fixe six motifs de dérogation. Dans la mesure où toutes ces dérogations semblent déjà transcrites dans notre droit dans les articles relatifs aux espèces protégées et à la régulation des espèces, je ne comprends pas quelle serait la plus-value apportée par le présent article. En effet, il est déjà possible aujourd'hui de prévoir des prélèvements d'oiseaux migrateurs causant des dégâts. J'ai ainsi souhaité interroger de nouveau le président de la Fédération nationale des chasseurs sur ce sujet dans le cadre d'un courrier que je lui ai adressé. Je l'avais d'ailleurs entendu en audition, tout comme le représentant de la Ligue Ma seconde réserve porte sur la justification du présent article au sein du présent projet de loi qui entend supprimer des surtranspositions pesant de manière injustifiée sur nos entreprises.

article transpose en droit interne la dérogation prévue à l'article 9 de la directive Oiseaux, qui permet de chasser des oiseaux migrateurs dans le but de prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux aux pêcheries et aux eaux lorsqu'il n'existe aucune solution satisfaisante. Cette dérogation est strictement conforme au droit de l'Union, dont elle se borne simplement à reprendre les termes J'insiste sur le fait qu'en tant que telle, elle n'introduit nullement un droit automatique de chasser ces espèces migratoires. Elle se borne à permettre qu'une telle dérogation soit autorisée à l'avenir sur la base d'un texte spécifique, sous réserve que les conditions prévues par la directive soient remplies, à savoir, premièrement, que des dégâts importants aux cultures soient constatés, qu'aucune autre solution satisfaisante ne permette d'y remédier, et troisièmement, qu'une telle mesure soit compatible avec le maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées. Cette dernière condition sera appréciée par un conseil scientifique qui va être mis en place pour éclairer les décisions de l'État. Le respect de ces conditions sera d'ailleurs contrôlé le cas échéant par le juge administratif. Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette mesure, qui ne porte en aucun cas atteinte à la protection des espèces migratrices. Elle se borne simplement à reprendre une faculté de dérogation dont le Gouvernement estime qu'il y a lieu de l'inscrire en droit interne dans le contexte de la mise en oeuvre d'une gestion adaptative des espèces chassables telle qu'annoncée à l'issue des discussions qui ont été conduites- et suivies de près au Sénat -, aussi bien avec les chasseurs qu'avec les associations protectrices de la nature. Cette nouvelle approche rend donc nécessaire de disposer de mesures permettant d'accroître la régulation des espèces qui causent des dégâts excessifs. Inversement, les espèces vulnérables vont faire l'objet de mesures accrues de protection.

Si on interdisait la chasse des oiseaux migrateurs et du gibier d'eau, la moitié des zones humides françaises disparaîtrait, car ce sont les chasseurs qui les entretiennent à grands frais

un signe ! Je ne suis pas nostalgique, mais je regarde le monde tel qu'il évolue, et je pense qu'il est temps de prendre des mesures de protection. C'est pourquoi je voterai ces amendements. La

pour pouvoir déterminer des quotas de prélèvement. Cette gestion adaptative consiste à redéfinir cycliquement la gestion d'une espèce et de son écosystème et constitue en elle-même une démarche scientifique qui nécessite de comparer continuellement les résultats des mesures de gestion aux données de terrain constatées, afin d'ajuster progressivement lesdites mesures.

pendant leur période de migration pour les chasses traditionnelles prélevant de petites quantités de spécimens, au motif de dégâts causés aux cultures, au bétail, aux pêcheries et aux eaux.

qui permet de déroger à l'interdiction de chasser édictée par transposition de la directive Oiseaux de 2009 pour prévenir des dommages agricoles, en introduisant les autres motifs de la dérogation prévue par cette directive. Ces motifs complémentaires n'ont pas été inscrits dans le projet de loi du Gouvernement, car ils ne répondent à aucun besoin, d'autres outils juridiques existant peut citer, par exemple, l'article L. 427-6 du code de l'environnement qui permet aux préfets d'organiser ponctuellement des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques pour des raisons de santé, de sécurité publique ou de conservation de la faune- un motif pour lequel le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir la possibilité du recours à la chasse.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande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

« les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai » ... Il y a pourtant une urgence impérative à obtenir, avec l'aide des agences de l'eau, dont les moyens doivent absolument être maintenus, une bonne qualité de la masse d'eau. aujourd'hui au regard de cet objectif prioritaire pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. À l'heure où la directive-cadre sur l'eau est en cours de révision, notamment pour aller plus loin dans le droit d'accès de tous à ce bien de première nécessité, nous estimons qu'il n'y a pas d'urgence à légiférer, surtout pour laisser entendre que, dans certains endroits, les pollutions pourraient continuer

Cet amendement vise également à supprimer l'article repoussant les échéances permises par la directive-cadre sur l'eau pour atteindre un bon état écologique des masses d'eau. Nous n'avons déjà

absolue, le report des échéances du fait des conditions naturelles risque d'avoir un effet démobilisateur sur les acteurs, à qui elle adresse, encore une fois, un signal très négatif.

De plus, cette disposition ne pouvant être prise en compte que dans les futurs schémas d'aménagement de la gestion des eaux pour la période 2022-2027, il serait souhaitable d'attendre au moins les conclusions des discussions européennes actuelles sur le projet de révision de la directive-cadre sur l'eau.

technique, la mesure se justifie pleinement sur le fond. En effet, certaines masses d'eau, du fait de leurs conditions naturelles, mettent beaucoup de temps à évoluer, quelles que soient les actions engagées pour les améliorer. Ce report ne pourrait ainsi concerner que quelques masses d'eau qui, pour des raisons indépendantes de la volonté des acteurs, sont plus lentes à se modifier. Au final, cela permet de ne pas démobiliser les acteurs en leur fixant des

échéance. Le présent article transpose certaines des dérogations prévues à ce titre qui n'ont pas été intégrées en droit interne. Il permet de reporter cette échéance,

La première dérogation, qui ne joue que dans le cas où les conditions naturelles elles-mêmes ne permettent pas d'atteindre les objectifs établis par la directive, reste très encadrée. Les conditions naturelles s'entendent en effet comme des conditions objectives, c'est-à-dire des conditions physiques ne permettant pas d'atteindre le bon état de l'eau dans un délai donné. Il s'agira, par exemple, du temps nécessaire à la résorption dans l'eau d'une substance dont l'usage est désormais interdit. De plus, cette dérogation ne pourra jouer que lorsque toutes les mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux auront été mises en oeuvre. La Commission a pris soin de le rappeler dans une note qu'elle a transmise au directeur de l'eau en décembre 2017.

Enfin, aucune régression de l'état des masses d'eau n'est autorisée. Le report du délai n'est possible que si l'état de la masse d'eau ne se détériore pas davantage. Les échéances pour mener les actions nécessaires au bon état des eaux ne sont donc pas modifiées, et cette disposition n'aura pas d'effet démobilisateur sur les acteurs concernés. S'agissant de Mayotte, il est justifié que ce territoire puisse bénéficier de toutes les dérogations que lui ouvre le droit européen en raison de son statut de région ultrapériphérique de l'Union. Dans

s'agissant, notamment, de la gestion de la pollution de l'air par les navires ou de la maîtrise du développement des éoliennes en mer. Il s'agit en effet d'enjeux essentiels. Rappelons qu'un navire de transport marchand cause autant de pollution aux particules ultrafines qu'un million de voitures. Les bateaux de croisière ne sont pas en reste ; or ce marché est en plein boom, avec une croissance à deux chiffres. On peut donc légitimement se demander quel sera l'effet de la suppression de cette mention sur cet aspect de la protection des milieux marins. Nous avons été alertés par des ONG environnementales, qui s'inquiètent profondément de cette suppression. De plus, la notion d'espace aérien surjacent est apparue dans la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, et on peut par conséquent considérer qu'il s'agit d'une surtransposition assumée correspondant à la volonté de mettre en lumière la nécessité de protéger les milieux marins dans leur globalité. La simplification ne doit pas être un prétexte pour une protection au rabais de notre environnement.

de la définition des eaux marines, et donc du champ d'application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. En effet, cette notion, insérée sur l'initiative du législateur, n'est pas conforme à la directive européenne et n'est, de fait, pas reprise par la stratégie nationale, elle-même publiée par décret. Cela n'empêche pas celle-ci pour autant de traiter indirectement de cet espace à travers des thématiques comme l'énergie éolienne, la pollution atmosphérique des navires, la protection des oiseaux, ou encore les pollutions lumineuses. Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable

L'article 18 supprime l'espace aérien surjacent du champ d'application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette inclusion constitue une surtransposition, dans la mesure où la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ne prévoit pas que les eaux marines, qui constituent le champ d'application de cette stratégie, incluent l'espace aérien surjacent. Cette surtransposition est dépourvue de tout effet pratique, faute d'avoir conduit à l'application de mesures à l'espace aérien dans le cadre de la stratégie marine adoptée par le décret du 23 février 2017. Elle est donc simplement une source éventuelle de confusion et de complexité. La disposition proposée à l'article 18 garantit la bonne cohérence du droit avec le droit de l'Union européenne et une meilleure sécurité juridique. Elle sera sans effet sur la protection de l'environnement, et ne modifie pas la stratégie pour la mer et le littoral. C'est pour cette raison que le Gouvernement est défavorable à cet amendement

Je tiens d'abord à préciser que nous ne sommes en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Néanmoins, nous nous interrogeons sur la pertinence de légiférer dans le domaine ferroviaire, alors que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été adoptée en juin dernier. Cette loi a profondément bouleversé feu notre Société nationale des chemins de fer français et ses agents. Certains des sujets sont traités dans le cadre des ordonnances prises en application de ladite loi et

Par ailleurs, les réseaux urbains et suburbains devraient être au coeur du projet de loi d'orientation des mobilités, qui prévoit une réforme globale de la gouvernance des mobilités.

Cet amendement vise à supprimer l'article excluant certaines portions du réseau ferroviaire du champ d'application des règles de gestion des installations de service. Pour ses auteurs, cette démarche de simplification, qu'ils soutiennent par ailleurs, aurait dû avoir lieu dans le cadre de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire ou des ordonnances qu'elle prévoit. Je suis d'accord, il aurait été plus pertinent de traiter l'ensemble de ces questions en une seule fois, mais cela ne me semble pas justifier le rejet complet de ces mesures, qui vont dans le sens souhaité d'une amélioration de la compétitivité des opérateurs ferroviaires

de l'amendement, la modification du code des transports proposée par le Gouvernement vise à introduire des dérogations qui n'étaient pas prises en compte jusqu'ici, alors qu'elles étaient permises par la directive 2012/34/UE, notamment concernant les obligations applicables aux installations de service. Ces simplifications sont susceptibles de bénéficier à des entreprises ferroviaires qui exploitent des services de transport de voyageurs en milieu urbain ou suburbain, ou à des opérateurs de proximité qui circulent hors du réseau ferré national. Dès lors qu'elles visent à prendre en compte l'ensemble de ces possibilités offertes par les directives européennes, ces dispositions ont leur place dans le projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions. Elles ne seront, par conséquent, pas traitées dans le cadre des dispositions à venir des ordonnances destinées à mettre en oeuvre la loi

Dans cette loterie des surtranspositions, je n'ai pas bien compris pourquoi ces articles nous sont soumis maintenant. Mme la rapporteur vient de rappeler qu'effectivement nous sommes

de manière très didactique, les causes de surtransposition. Il a évoqué des délais trop précipités, des textes trop techniques- à l'échelon européen, les directives sont issues de négociations longues et complexes -, et donc les risques de confusion

Le présent article prévoit d'exempter certaines entreprises ferroviaires- on aimerait bien nommément savoir lesquelles -de l'obligation de séparation comptable de leurs activités de gestion d'infrastructures et de services de transports ferroviaires. Il vise introduire une simplification pour des entreprises ferroviaires de voyageurs ou de marchandises qui n'exploitent que des services suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes utilisant une infrastructure ferroviaire. Comme vous le constatez, c'est assez pointu. Il s'agit en l'occurrence d'entreprises qui opèrent sur des lignes spécifiques, comme des lignes touristiques ou des lignes dédiées à des opérateurs de fret ferroviaire de proximité. Comme nous l'avons déjà souligné, nous ne sommes en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs, mais certains termes utilisés dans ce texte, comme la notion de réseaux locaux ou régionaux autonomes, constituent pour nous réellement

Cependant, cet argument ne me semble pas de nature à justifier la suppression de cette disposition, qui reprend une exclusion stricte du champ d'application de la directive, d'autant que le ministère m'a fourni des indications sur les portions de réseaux qui pourraient être concernées. Je les ai d'ailleurs fait figurer dans mon rapport. Il s'agit en Il s'agit en outre de transposer en droit interne une exclusion stricte du champ d'application de la directive. Ce n'est pas une possibilité de dérogation laissée à la discrétion des États membres. La commission spéciale a émis un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? La rédaction

permis par la directive 2012/34/UE. La notion de réseaux locaux ou régionaux autonomes n'est certes pas définie par la directive ni en droit national, mais cette incertitude sur ses contours correspond à la marge d'appréciation laissée aux États membres, afin de permettre la mise en oeuvre la plus pragmatique possible. La disposition proposée introduit une simplification qui peut profiter potentiellement aux opérateurs de proximité. Elle trouve sa place dans le cadre d'un texte à supprimer les surtranspositions, dans la mesure où elle permet de prendre en compte toutes les flexibilités autorisées par la directive 2012/34/UE. Une telle disposition ne pourrait pas être introduite dans les ordonnances « ferroviaires » qui seront prises en application de la loi du 27 juin 2018

que la France s'est engagée- toutes les majorités successives sont donc comptables de cet engagement -dans un système de mise en concurrence des transports ferroviaires reposant sur le principe que le gestionnaire du réseau, c'est-à-dire des rails, de l'infrastructure, et les transporteurs sont différenciés. Toute l'Europe, souvent de façon très laborieuse, a appliqué progressivement cette différenciation. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire que nous avons adoptée n'est que le cinquième ou sixième exercice législatif français destiné à mettre en oeuvre cette séparation. On a juste mis vingt ans à s'apercevoir qu'il y avait quelques fragments de réseau pour lesquels cette séparation de l'exploitant du transport et du gestionnaire du réseau n'avait pas de sens, car il n'y avait qu'un seul exploitant sur un réseau limité.

le Conseil d'État lui-même a remarqué que cette qualification de réseau autonome était insuffisante pour bien distinguer les parties de réseau et ne pas risquer de déliter le réseau ferroviaire national. S'il s'agit, pour faire simple, de faire plaisir à quelques entreprises

réseau. Il faut un maximum d'efficacité sur ce réseau, et qu'il soit « circulé » entièrement et complètement. Si certaines parties bénéficient de règles différentes, c'est une source de problèmes importants.

de l'obligation d'être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire. On retombe sur cette problématique que je viens d'évoquer au sujet du qualificatif « autonomes », qui est insuffisamment précis et qui pourrait entraîner des confusions.

toutes les dérogations relatives à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire permises par la directive 2012/34/UE. Il rentre ainsi entièrement dans le cadre du projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions. la notion de réseaux locaux ou régionaux autonomes n'est certes pas définie par la directive ni en droit national, mais cette incertitude sur ses contours correspond à la marge d'appréciation qui est précisément laissée aux États membres pour permettre la mise en oeuvre la plus pragmatique et la plus proche du contexte local et national possible. La mesure proposée introduit une simplification qui peut profiter potentiellement aux opérateurs de proximité. Par ailleurs, une telle disposition ne pourrait pas être introduite dans les ordonnances « ferroviaires » qui seront prises en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, dans la mesure où les habilitations que cette dernière contient ne permettent pas de revenir sur une ancienne transposition. Il faut noter que la suppression de l'obligation de détenir une licence d'entreprise ferroviaire n'aura pas d'impact sur la sécurité ferroviaire, celle-ci visant en premier lieu à s'assurer de la bonne santé financière des entreprises ferroviaires et de l'honorabilité de ses dirigeants.

L'article 22 durcit les conditions de mise à disposition des installations de service non utilisées. Le domaine traité par cet article a fait l'objet de débats lors de l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire par le Parlement. Les ordonnances autorisées par ce texte sont en cours de finalisation et risquent donc d'interférer avec les dispositions du présent projet de loi

Quel est l'avis de la commission spéciale ? Pour les mêmes raisons que précédemment, et même si je comprends les réserves des auteurs de l'amendement sur la méthode, l'avis de

Une telle disposition, qui vise à prendre en compte toutes les possibilités offertes par la directive 2012/34/UE, a vocation à être introduite dans le présent projet de loi. les surtranspositions. Elle n'aurait, en tout état de cause, pas pu être intégrée aux projets d'ordonnance qui devront être pris aux fins de la mise en oeuvre de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. En effet, les articles d'habilitation que celle-ci contient ne permettent pas

Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d'entreprises ferroviaires qui opèrent sur des réseaux « séparés sur le plan fonctionnel du reste du réseau et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs- j'insiste sur le mot « voyageurs » -ou de marchandises ». Il supprime, pour certains conducteurs des trains concernés, l'obligation d'être titulaires d'une licence ferroviaire. La licence ferroviaire ne serait donc plus nécessaire. N'est-ce pas une sorte de permis de conduire ? La licence pour conduire un train peut-elle être optionnelle, car on parle bien de voyageurs ? Pour obtenir cette licence, il faut satisfaire à certaines conditions de formation, de connaissances professionnelles. Il faut également justifier d'aptitudes physiques et psychologiques. Ladite licence est associée, la plupart du temps, à des attestations délivrées par un exploitant ferroviaire. Elle est en outre précisément destinée à harmoniser la certification entre les États membres de l'Union européenne. Nous sommes pour le moins dubitatifs. N'y a-t-il pas, de toute évidence, une question de pure sécurité ? Oui, car il est bien question ici de simplification de règles de sécurité, et ce, je n'ose l'ajouter, pour des raisons financières.

22 000 euros Nous nous opposons à cette vision purement comptable. La réduction des coûts ne peut en aucun cas justifier de prendre des risques avec la sécurité pour les opérateurs ferroviaires et les usagers de ces transports. Sans autre précision ni garantie, nous considérons que cette suppression de l'exigence de certification n'est pas une bonne nouvelle pour la sécurité ferroviaire. Nous demandons, à l'inverse, un haut niveau d'exigence pour l'ensemble des conducteurs de train à l'échelon européen. Nous ne supportons plus ce nivellement qui tend toujours vers le bas et le moins-disant social, alors que les enjeux d'une Europe ferroviaire sûre, fiable et performante sont d'une actualité criante, au moment même où le train apparaît comme un levier pertinent et incontournable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre

de l'obligation de détenir une licence. Je comprends et partage les préoccupations liées à la sécurité que viennent d'exprimer les auteurs de ces amendements. Je me suis personnellement assurée de deux points

aux entreprises concernées ; je pense, par exemple, à l'obligation d'élaborer des systèmes de gestion de la sécurité qui doivent permettre de maintenir le niveau de sécurité requis pour

Une telle disposition, qui vise à prendre en compte toutes les possibilités offertes par la directive 2007/59/CE, a vocation à être introduite dans le projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions.

4, 10, 13, 24, 25, 26 et 27, qui font l'objet de la procédure de législation en commission.

de la totalité des surtranspositions en droit français des directives européennes est, une fois de plus, l'agriculture. Oui, une fois de plus, madame la secrétaire d'État, rien n'a été dit sur toutes les problématiques que nous connaissons. Rien sur l'application du droit à l'erreur dans le cadre de la PAC.

nous en avons encore ajouté une couche avec la loi ÉGALIM, ce qui explique peut-être pourquoi le Gouvernement n'a rien proposé sur l'agriculture. Je vous le rappelle, nous avons surtransposé à outrance avec l'interdiction des remises-rabais-ristournes, la séparation capitalistique, les plastiques alimentaires,

en particulier en matière de droit de la consommation, en matière environnementale ou en matière de sécurité, comme on vient de le voir.

D'une manière générale, comme je l'ai dit au début de mon propos, il y a un vrai problème de méthode dans le choix des surtranspositions. Surtout, on ne voit pas la cohérence d'ensemble sur le choix des thématiques, sur l'équilibre entre elles au regard de ce qui est recherché, c'est-à-dire la simplification. Le débat a été très révélateur sur ce plan. Sur nombre d'articles, on a dit comprendre

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, mes chers collègues, à l'issue de nos travaux sur ce projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, je tiens à féliciter le Sénat d'avoir joué depuis plusieurs mois un rôle moteur dans l'identification de cet enjeu. faut toutefois, mes chers collègues, faire preuve d'une volonté claire de supprimer les surtranspositions et de nous attaquer de front aux contraintes les plus coûteuses pour nos entreprises. Il ne faut pas nous contenter de mesures anecdotiques

pourrait citer des exemples parlants. Je vous adresserai quelques mots pour le futur. Nous n'avons pas pu- nous l'avons souligné à de nombreuses reprises -aller aussi loin que nous l'aurions souhaité dans la dé-surtransposition, nous trouvant limités par le champ du texte. Notre assemblée examinera dans les prochains mois des textes de grande importance- projet de loi Mobilités, projet de loi PACTE, par exemple ... Je vous invite, pour poursuivre le travail modestement entamé aujourd'hui, à rester vigilants sur l'impact des mesures votées dans cet hémicycle. Il faut systématiquement nous interroger sur les conséquences concrètes de nos propositions législatives et de nos amendements : pour qui créent-ils des coûts et des contraintes ? Instaurons-nous délibérément des obstacles à la compétitivité de nos entreprises et provoquons-nous une surcharge de travail pour nos administrations ? À l'inverse, il ne faut pas hésiter à proposer de nouvelles suppressions de surtranspositions dès qu'un texte en offre l'opportunité. Ainsi, le projet de loi PACTE procédera à la ratification de vingt-trois ordonnances de transposition de directives. Pour que le travail réalisé lors de l'examen du présent projet de loi puisse réellement payer, il nous reviendra de contrôler ensemble les travaux ultérieurs du Gouvernement et de ne pas instaurer nous-mêmes de nouvelles surtranspositions. La parole Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au terme de nos travaux, je tiens, en ma qualité de président de la commission spéciale, à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la rédaction, à l'examen et, au final, à l'adoption de ce texte. Je remercie en particulier les deux rapporteurs, M. Cadic et Mme de Cidrac, ainsi que nos équipes, qui ont fait un travail considérable. L'exercice auquel nous nous sommes livrés est nouveau dans la mesure où, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un texte législatif est consacré à la suppression de surtranspositions, suppressions ondoyantes, diverses et manifestement, pour certains de nos collègues, quelquefois déroutantes ! L'essentiel, c'est que notre assemblée vient de supprimer vingt-trois surtranspositions- si j'ai bien compté ce qui nous encourage à continuer dans cette voie, en liaison avec le Gouvernement. En effet, il ne suffit pas de s'en prendre aux trop nombreuses et trop contraignantes normes, surtranspositions ... Encore faut-il diminuer leur nombre et éviter d'en créer de nouvelles ! Telles sont les raisons pour lesquelles nous discuterons prochainement de ma proposition de résolution et ultérieurement d'une proposition de loi. Quant à la commission des affaires européennes, elle remplira prochainement pleinement le rôle qui lui est assigné par le Sénat, un rôle d'alerte en cas de risque de surtranspositions de directives ou de règlements européens. Voici quel sera